J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur la proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Par lettre en date du 19 décembre, M. Didier Guillaume, président du groupe socialiste et républicain, demande l'inscription à l'ordre du jour réservé à son groupe du jeudi 1 février 2018 -de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, présentée par Mme Nicole Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain -et de la proposition de loi relative à la réforme de la caisse des Français de l'étranger, présentée par MM. Jean-Yves Leconte, Richard Yung, Mmes Claudine Lepage et Hélène Conway-Mouret. Acte est donné de cette demande. L'ordre du jour appelle l'examen de quatre projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. commission, l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet

Parmi les divergences majeures qui ont persisté entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative, j'insisterai sur deux dispositions qui, à elles seules, peuvent justifier l'échec de la commission mixte paritaire. La première, qui aurait pu suffire à empêcher un accord, concerne le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. L'opposition que votre assemblée a manifestée sur ce sujet vous a conduits à rejeter en bloc les mesures qui concourent à la mise en oeuvre du dispositif. Une nouvelle fois, le Sénat a privilégié la mise en place d'un prélèvement mensualisé assis sur les revenus de l'année, dispositif dont une mission de l'Inspection générale des finances a explicitement identifié les limites. Le rapport remis au Parlement concernant l'analyse des options alternatives à la mise en place du prélèvement à la source indique par ailleurs et de manière claire que la substitution à la retenue à la source sur les salaires d'un prélèvement calculé par l'administration fiscale sur la base des dernières données transmises par les payeurs de revenus constituerait une solution « dégradée » au regard des bénéfices attendus pour le contribuable. un tel prélèvement mensualisé n'offrirait pas tous les avantages que procure, selon le Gouvernement, un prélèvement s'adaptant chaque mois aux revenus versés, de façon immédiate et automatique.

En définitive, vous aurez compris que, sur ce point, le Gouvernement et la majorité présidentielle assument clairement le choix qui est le leur d'un véritable prélèvement à la source pour nos concitoyens, avec tous les bénéfices qu'il comporte. La seconde divergence majeure que je veux souligner concerne très directement le solde budgétaire de l'État, qu'un certain nombre de dispositions adoptées par votre assemblée concourent à dégrader, par la réduction des recettes et l'augmentation des dépenses.

En ce qui concerne l'augmentation des dépenses, vous avez adopté, entre autres mesures, la suppression d'un prélèvement de 27 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence française pour la biodiversité et modifié les plafonds d'affectation d'un certain nombre de taxes.

pense en particulier à l'extension des mesures en faveur de la libération du foncier à la zone B1, par l'application d'un coefficient de densité de 80 %, au lieu de 90 %, et l'ajout d'une évaluation avant le 1 septembre 2020.

normal ! D'abord, l'Assemblée nationale a confirmé, sans surprise, la mise en oeuvre du prélèvement à la source au 1janvier 2019. Nous considérons toujours qu'il pénalisera des contribuables, notamment ceux qui bénéficient

On aurait pu s'entendre, car nous n'étions pas opposés à une évolution du système ; mais l'Assemblée nationale a rejeté la proposition alternative du Sénat, consistant à mettre en place un prélèvement contemporain et mensualisé sur le revenu, opéré par l'administration fiscale.

la commission des finances avait adopté un amendement avec avis favorable du rapporteur général, mais le Gouvernement s'est opposé à la mesure cette nuit. Il faut croire que la copie du Gouvernement était parfaite ... Parfaite ! ... et qu'aucun aménagement ne pouvait y être apporté par les parlementaires

nous souhaitions- c'était également une position assez consensuelle du Sénat -que les plates-formes de réservation en ligne ne puissent plus verser le montant des loyers perçus sur des cartes anonymes prépayées à l'étranger, car, je le dis

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le vice-président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues,

Il faut reconnaître que les délais d'examen de ce dernier texte budgétaire de l'année sont serrés : fin de la première lecture vendredi dernier, réunion et échec de la commission mixte paritaire avant-hier, nouvelle lecture à l'Assemblée nationale cette nuit vers deux le tout en alternance avec l'examen des autres textes. Chaque année, nous déplorons cette organisation de nos travaux, mais chaque année rien ne change, malheureusement ... Lors de la réunion de la commission des finances de ce matin, nous avons constaté, sans surprise, le rétablissement de la plupart des dispositions du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, en particulier sur le prélèvement à la source, qui est la réforme majeure de ce texte. S'il n'y a pas vraiment lieu de s'étonner de ce retour au texte initial, on peut tout de même regretter la suppression de certaines modifications du Sénat, comme l'interdiction des cartes prépayées sur les plates-formes en ligne et d'autres mesures sur la fiscalité du numérique, qui constituaient des avancées et visaient à lutter contre la fraude. Il faudra nécessairement avancer sur ces questions un jour ou l'autre, le législateur ne pouvant indéfiniment rester en retard sur les mutations technologiques et les nouveaux usages qu'elles engendrent. Pour le reste, la soixantaine d'articles encore en discussion portent sur des mesures extrêmement variées et techniques, qui n'appellent pas de remarques particulières et méritent d'être adoptées en l'état.

Je ne doute pas que cette décision sera appréciée sur le terrain, en particulier dans le Lot, la Gironde et les Hautes-Pyrénées, ma chère collègue Carrère, qui abritent de magnifiques parcs zoologiques participant à leur façon à l'attractivité de nos territoires. La mise en place du prélèvement à la source, qui paraît désormais inéluctable, continue de susciter des débats. La majorité sénatoriale a proposé une mesure plus limitée : le prélèvement contemporain, qui consiste à améliorer le système existant sans en bouleverser les fondements, si complexes. Si la majorité de mon groupe est plutôt favorable à cette réforme, soutenue par une majorité de Français, nous serons attentifs à sa mise en oeuvre concrète.

Sur toutes les travées, nous constatons, en tant qu'acteurs de terrain, les dégâts de la désertification des territoires ruraux et des villes moyennes. Nous ne voulons pas que se creuse l'écart entre une France pourvue de tous les atouts pour son développement et une autre fragilisée, parfois délaissée par les pouvoirs publics. C'est aussi la voix de nos concitoyens qui se sentent relégués que nous portons dans cet hémicycle. Je ne doute pas, monsieur le secrétaire d'État, que vous serez sensible à la nécessité de donner à nos collectivités territoriales les moyens financiers de faire vivre le principe républicain d'égalité. Nous y serons très sensibles. En conclusion,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mes chers collègues, je pense avoir identifié le point qui, au moins à ce stade du constat, est susceptible de nous mettre d'accord : la procédure budgétaire dans son épure actuelle est à bout de souffle. Ce collectif budgétaire de fin d'année en est l'illustration : un examen au pas de charge, une inflation du nombre d'articles du fait de l'ajout d'amendements, notamment gouvernementaux mais pas uniquement, dans chaque assemblée et, au bout du compte, l'équivalent législatif d'un ancien magasin du Pont Neuf ... On y trouve de tout Mais, en réalité, nous ne nous y retrouvons plus, et cela sur toutes les travées. Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a pris l'engagement devant nous- cela ne manque pas de courage -de ne plus prendre de décrets d'avance au mois de novembre et de faire du collectif de fin d'année un texte purement technique. Cet engagement est totalement en cohérence avec l'exigence de sincérité du Gouvernement sur la loi de finances initiale et, plus largement, sur les textes financiers, une exigence qu'il s'emploie à respecter depuis juillet dernier. Nous aurons un rendez-vous constitutionnel en 2018, qui sera une fenêtre d'opportunité pour améliorer les conditions de travail du Parlement. Dix ans après la réforme dite « Sarkozy », qui a comporté des avancées, le compte n'y est toujours pas, comme l'attestent les nombreux appels publics à réformer les modalités d'examen de la loi de finances. Le diagnostic est largement partagé. Les députés avancent ainsi une proposition bienvenue de rééquilibrage du temps d'examen des textes financiers, aujourd'hui concentré sur le temps de la prévision et de l'autorisation, mais réduit pour le volet de l'évaluation et du contrôle de l'exécution. À droit constant, il serait par exemple souhaitable de consolider la discussion du volet recettes du projet de loi de finances et du projet de loi Il est paradoxal d'avoir une approche « toutes administrations publiques », mais une dispersion entre plusieurs textes ! Il ne serait d'ailleurs pas incohérent de discuter également des articles non rattachés- en simplifiant, les crédits d'impôt -en amont de la seconde partie. Je me permets un aparté : si nous, au Sénat, souhaitions contribuer, comme c'est notre rôle, à la création d'une nouvelle catégorie de lois de finances, consacrées aux finances locales, il faudrait que nous veillions à la fois aux contraintes de temps- quand discuter ? -et, bien entendu, de champ- que discuter S'agissant de la seconde partie, on pourra se demander s'il est de bonne politique d'avoir autant de rapporteurs spéciaux et de rapporteurs pour avis sur les différentes missions budgétaires. Pardonnez-moi cette observation qui est un peu celle d'un Huron au palais du Luxembourg, mais j'ai souvent pensé à la formule, fameuse, d'Edgar Faure : « litanie, liturgie, léthargie » pendant les débats en séance publique, après de riches débats et de nombreuses auditions très intéressantes en commission. À tous les stades de la procédure- mais sans doute est-ce chimérique il serait probablement plus raisonnable pour le Gouvernement de ne plus déposer des amendements hors délai, ou alors de fournir systématiquement une étude d'impact. Le groupe La République En Marche avait eu l'occasion de s'exprimer en ce sens lors de l'examen en urgence du collectif « flash » faisant suite à la censure de la taxe de 3 % sur les dividendes. Le Parlement doit veiller à ce que les principaux amendements gouvernementaux en matière fiscale soient suffisamment documentés. Le rapporteur général, qui est plus chevronné que moi, l'a répété : nous ne pouvons plus légiférer à blanc, sans un minimum de travail en commission des finances. Faut-il confier l'examen du budget à des algorithmes ? Pas encore. Car des pistes stimulantes ont été avancées, pas uniquement au Palais-Bourbon, mais aussi dans certains. Ainsi, nous pouvons consacrer davantage de temps au contrôle de l'exécution des lois de finances. Les lois de règlement, en dépit des ambitions initiales de la LOLF, sont devenues, ou plutôt sont restées, des astres morts. Comment prétendre vouloir améliorer la loi fiscale quand on ne prend jamais véritablement le temps d'en évaluer les effets ?

En dopant ce volet de l'évaluation des dépenses publiques, le Parlement aura un rôle substantiel en matière de contrôle, mais aussi une meilleure connaissance de la construction budgétaire proposée par le Gouvernement. Nous avons la chance de bénéficier de l'assistance précieuse de la Cour des comptes pour nos travaux de contrôle et d'évaluation. Je suis plus réservé sur l'idée, récurrente, d'une intégration de la Cour des comptes comme institution à part entière du Parlement, compte tenu de ses activités juridictionnelles. Nous pourrions également renforcer nos liens avec d'autres organismes menant un travail d'évaluation qui mérite d'être porté dans le débat public- je pense à la Banque de France et à l'INSEE le cas échéant à travers une politique un peu volontariste en matière de mobilités. Nous avons ici d'excellents juristes ; attirer dans ses murs des économistes et des statisticiens pourrait être pertinent. Il nous faut veiller aussi à enrichir davantage nos travaux d'évaluation des recherches universitaires en matière économique : de Philippe Aghion à Gabriel Zucman, en passant par Jean Tirole et Thomas Piketty, nous avons la chance d'avoir des têtes chercheuses en France, et il serait positif de les associer davantage à nos travaux.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ainsi donc, comme pour la loi de finances pour 2018, tout en étant d'accord sur les trois quarts du texte, la majorité sénatoriale n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la majorité de l'Assemblée nationale, alors même que les uns et les autres défendent globalement les mêmes intérêts. Des questions de positionnement politique en sont sans doute la rançon.

80 % des Français ne payaient,, que 16 à 17 % de l'impôt sur le revenu- en tout cas, de l'impôt progressif. La majorité de cet hémicycle juge cette situation anormale et propose donc un ensemble de mesures d'allégement d'impôt touchant, au fil des amendements, aux impôts immobiliers, à l'activité des professions libérales, aux revenus de capitaux mobiliers, à l'impôt sur les sociétés ou encore aux droits de mutation. Ce que ne dit pas la droite sénatoriale, c'est que ceux qui échappent pour tout ou partie à l'impôt sur le revenu subissent les 150 milliards d'euros de TVA, les 130 milliards d'euros et les 40 ou 50 milliards d'euros de la fiscalité écologique, sans parler des droits sur le tabac, les alcools et les sodas, entre autres exemples. Ces 80 % qui ne sont pas redevables, partiellement ou totalement, de l'impôt sur le revenu sont aussi ceux qui vivent dans les quartiers populaires, dans nos cantons ruraux enclavés et dans les grandes villes soumises à la pression spéculative, là où le service public d'État est de plus en plus défaillant et rendu incapable de maintenir le lien social. Jean Jaurès a dit que « le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Une maxime toujours d'actualité ! Il y a peu de temps encore, j'étais maire d'une de ces communes populaires où vivent des salariés, des familles, des ouvriers, des retraités, des gens modestes qui font clairement partie de ces 80 % que vous voudriez imposer plus encore. Songez-y : le tiers des habitants de ma commune a déclaré en 2016 un revenu imposable inférieur à 10 000 euros

n'est que ses auteurs ont beaucoup manié le décret d'avance et d'annulation des crédits. Cet exercice budgétaire restera marqué par quelques faits essentiels. retiendra la sous-budgétisation des contrats dits « aidés ». Cette situation a créé un émoi légitime lors de la rentrée scolaire 2017-2018,

L'ouverture de nouveaux contrats pour la rentrée ne doit pas faire oublier l'essentiel dans cette affaire. Pourquoi tant de collectivités locales et/ou d'associations se voient-elles dans l'obligation de passer par ce type de contrats pour disposer de personnels qui travaillent au contact direct du public ? Par voie de conséquence, ne serait-il pas temps de passer de la gestion de contrats aidés à l'insertion professionnelle réelle, singulièrement par la voie des concours normaux de la fonction publique ? Là où il faut recruter, surtout quand ces recrutements sont nécessaires à l'intérêt général, recrutons !

Pour le reste, la situation sociale s'est suffisamment détériorée dans notre pays pour que le budget de l'État ait encore été sollicité, par exemple, pour financer l'allocation aux adultes handicapés. Du côté des ouvertures de crédits, il nous faut quand même évoquer le problème de la croissance continue, au fil des années, des dépenses liées aux opérations militaires extérieures, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la présence de nos troupes notamment au Mali, en Syrie, en Centrafrique ou en Afghanistan. Sans Sans débattre du bien-fondé de telle ou telle intervention, je crois, tout comme les membres de mon groupe, que la France devrait faire autre chose au-delà de ses frontières. Bien sûr ! Il est grand temps que la politique extérieure de notre pays fasse place au développement des pays du Sud que nous aidions véritablement ces pays à sortir des difficultés qu'ils connaissent. La jeunesse des pays dits « pauvres » est suffisamment riche de potentiels et d'idées pour que nous l'aidions à construire un avenir plus radieux pour eux, comme pour nous.

également la relation entre l'administration et le contribuable, pourtant fondamentale en l'état actuel des choses. Comment arguer de la plus grande efficacité de la retenue à la source, alors que l'impôt sur le revenu est recouvré à hauteur de 98 %, notamment au travers de la mensualisation ? Signalons que les fraudes constatées portent en général soit sur des revenus d'activité non salariée, soit sur des revenus d'origine étrangère. En outre, cela ne dispensera pas le contribuable de faire une déclaration de constatation en fin d'année

La volonté d'une plus grande transparence sur les finances publiques, le souci de sincérité et de crédibilité, notamment dans l'évaluation des hypothèses de croissance, sont autant de progrès que nous saluons. Après les errements du précédent gouvernement et la coûteuse insincérité du budget 2017, le changement de méthode est indéniable et mérite d'être souligné. Maintenue à 1,7 %, la prévision de croissance est prudente. Cette prévision est en deçà des récentes estimations publiées par la Commission européenne, l'OCDE et le FMI qui tablent tous sur une croissance de 1,8 % pour l'année 2017. Hier encore, l'INSEE relevait une nouvelle fois sa prévision de croissance pour 2017, la portant à 1,9 %, chiffre le plus haut depuis 2011. La prévision de déficit reste également inchangée à 2,9 % du PIB. Malgré cette apparente stabilité, le déficit pour 2018, initialement attendu à 2,6 %, sera finalement de 2,8 %. Cet écart s'explique principalement par les 5 milliards d'euros que va devoir supporter l'État dans le cadre du contentieux de la fameuse taxe à 3 % sur les dividendes. Monsieur le secrétaire d'État, qu'il nous soit permis ici de vous redire notre inquiétude. Dans ce dossier, les demandes de remboursements

La sortie de la France de la procédure de déficit excessif s'inscrit plus que jamais en pointillé. Cette fragilité budgétaire est d'autant plus préoccupante qu'une épée de Damoclès pèse au-dessus de nos têtes, en l'occurrence celle d'une remontée des taux d'intérêt, largement artificiels et anormalement bas aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous avons bénéficié d'un environnement économique favorable qui explique presque à lui seul la hausse des recettes de l'État dans ce second projet de loi de finances rectificative, soit un surplus de 2,1 milliards d'euros par rapport aux prévisions initiales. Le retour à une conjoncture propice explique que, dans ce texte, la prévision de recettes de TVA soit supérieure de 900 millions d'euros à ce qui était prévu. sur les produits énergétiques, la TICPE, dopées de 800 millions d'euros par rapport aux précédentes prévisions. La baisse de 1,5 milliard d'euros du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne masque, elle aussi, la réalité de l'embellie de nos finances publiques. Monsieur le secrétaire d'État, nous l'avons dit et le répétons aujourd'hui : des efforts doivent être fournis au niveau de la dépense publique qui, au lieu de 1,8 %, augmentera de 1,9 % en 2017. Pour assainir nos comptes publics, il nous faut commencer par maîtriser la dépense

Nombre d'entre eux l'avaient été à la hâte, sans examen préalable ni chiffrage. Nous avons regretté que le collectif budgétaire de fin d'année fasse de nouveau office de « texte-balai », avec des mesures dont l'objet a peu à voir avec la « rectification » de la loi de finances initiale. Nous avons surtout regretté qu'il ait fallu attendre l'ultime projet de budget pour que soient intégrées des dispositions aussi importantes que la liquidation de la société Ecomouv'ou la création du fonds d'urgence en faveur des départements, respectivement pour 339 millions d'euros et 100 millions d'euros. Est-ce acceptable ?

Au groupe Union Centriste, nous n'avons aucune hostilité de principe à l'égard de ce prélèvement. L'une des principales difficultés soulevées réside dans le modèle même de notre impôt sur le revenu.

La transformation des entreprises en collecteurs de l'impôt n'est pas le moindre des problèmes. C'est pourquoi nous avons soutenu la proposition du rapporteur général de la commission des finances, qui vise à y substituer un prélèvement mensualisé et contemporain qui, tout en conservant la suppression du décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt, déleste les entreprises du fardeau de la collecte. Comme il fallait s'y attendre, le texte voté cette nuit par l'Assemblée nationale a confirmé la mise en oeuvre du prélèvement à la source au 1janvier 2019. Il est néanmoins malheureux qu'aucune des modifications apportées par le Sénat n'ait prospéré à l'issue de la nouvelle lecture du texte à l'Assemblée nationale. Concernant certaines d'entre elles, il nous semble qu'un consensus aurait pu être trouvé.

Le récent scandale des cartes de crédits rechargeables proposées depuis Gibraltar par une célèbre plate-forme de location ne commande-t-elle pas une action rapide ? L'heure n'est plus à l'adaptation des plates-formes à la législation fiscale, mais à l'adaptation de la législation fiscale aux pratiques parfois frauduleuses de ces plates-formes. Au regard du sort presque certain qui attendrait les nouvelles propositions du Sénat, le groupe Union Centriste votera la motion tendant à opposer la question préalable déposée par le rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, que je tiens ici à féliciter pour la qualité de ses travaux. de vous remercier,

Voilà déjà une bonne nouvelle ! L'année 2017 se termine sur deux informations qui vont en sens contraire. L'une est positive : l'INSEE révise une nouvelle fois à la hausse le taux de croissance de l'année 2017, à 1,9 %.

que nous allons petit à petit. Cette année 2017 et la lecture rétrospective de nos travaux tout au long de la période budgétaire, avec une loi de programmation

parlerai pas de l'amendement gouvernemental sur la contractualisation, déposé en séance au Sénat au mépris de la règle constitutionnelle de l'entonnoir

est possible, susceptibles d'être intégrées et mieux entendues dans le cadre du projet de loi de finances. Sans doute, notre première expérience en la matière, qui portait sur le financement du logement social, n'a-t-elle pas été à ce totalement couronnée de succès. Évidemment, c'est un pur euphémisme ! Pour autant, c'est la voie que nous devons emprunter si nous voulons que la voix des élus de terrain que nous sommes soit mieux entendue et, je l'espère, mieux respectée à l'avenir,

commission des finances, mes chers collègues, nous examinons à nouveau le second projet de loi de finances rectificative pour 2017. La commission mixte paritaire a de nouveau échoué à réconcilier les positions des deux assemblées. Pourtant, les deux majorités se retrouvent sur la volonté de solder les comptes du précédent quinquennat C'est au moins un dénominateur commun qui aurait pu nous réunir dans le cadre du dernier collectif budgétaire de l'année. Pour mémoire, les biais de construction de la loi de finances initiale pour 2017 auront nécessité une ouverture de 6,2 milliards d'euros de crédits en cours d'exercice, un montant tout à fait inédit par son ampleur. De ce point de vue, nous ne pouvons que nous réjouir de voir que vous semblez avoir tiré les leçons de ces sous-budgétisations chroniques, L'Assemblée nationale a néanmoins rejeté avec méthode des mesures qui avaient fait consensus au Sénat, comme les mesures contre la fraude fiscale ou celles sur la fiscalité du numérique. Cette manière de faire nous interroge, alors que ces mesures apparaissent de bon sens et sont le fruit de travaux approfondis au sein de notre assemblée. Nous souscrivons aux remarques du rapporteur général sur la nécessité d'un plus grand respect des travaux du Sénat, lorsqu'ils vont manifestement dans le sens de l'intérêt général. Plus substantiellement, l'Assemblée nationale a refusé le prélèvement mensualisé et contemporain proposé par le Sénat, qui avait l'avantage de conserver la suppression du décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt, et un autre avantage de moins peser sur les entreprises. Si nous déplorons qu'un compromis entre ces deux visions n'ait pas pu être trouvé, notre groupe n'est pas, par principe, opposé au prélèvement à la source. Certes, ce type de réforme occasionne toujours des effets d'aubaine et des coûts afférents. Mais, si elle est bien menée, dans une logique de simplification et de bienveillance pour le contribuable et l'entreprise, elle peut contribuer à rendre notre système fiscal plus juste et plus efficace. L'idée du prélèvement à la source n'est d'ailleurs pas nouvelle et nous pourrions tirer avantage des expériences des pays voisins. Tous les grands pays d'Europe ont déjà opté pour le prélèvement à la source, l'Allemagne au premier chef. Néanmoins, l'amendement du Sénat avait le mérite de pointer du doigt plusieurs inconvénients de cette réforme : je pense aux interrogations portant sur la « familialisation » de l'impôt sur le revenu, les incertitudes concernant les crédits d'impôt existants ou encore les difficultés de mise en oeuvre pour les PME. Nous attendrons du Gouvernement qu'il prenne en compte les inquiétudes légitimes de notre assemblée et qu'il veille à mettre en oeuvre une mesure équilibrée et réaliste. Rien ne serait pire que la mise en place d'une « usine à gaz » lourde et complexe. Je voudrais maintenant revenir sur un point que nous avons abordé hier lors des discussions autour du projet de loi de finances. Le Sénat avait introduit dans ce second projet de loi de finances rectificative des amendements relatifs à l'aménagement de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, notamment en faveur des détenteurs de monuments historiques.

Hélas, nous sommes passés collectivement à côté de l'occasion d'améliorer l'IFI dans le cadre du projet de loi de finances, et cela n'est pas la faute de l'Assemblée nationale.

La France détient toujours le record européen de la dépense publique, de la pression fiscale et de la dette publique ! Mes chers collègues, en 2022, malgré les annonces, le différentiel d'endettement avec l'Allemagne sera sans précédent dans l'histoire récente. Ce simple fait devrait nous conduire à redoubler d'efforts. Derrière les chiffres et les pourcentages, il y va de notre influence politique en Europe et dans le monde. Nous sommes ici bien loin des calculs politiciens. Tout doit être tenté de courage de la part du Gouvernement, d'une part, et une approche constructive et pragmatique de la part de chacun d'entre nous sur cette question d'intérêt national,

un grand nombre de nos propositions devaient être reprises par les députés. Néanmoins, sous la pression du Gouvernement, tout a été balayé en séance ! Monsieur le secrétaire d'État, nous ne comprenons pas du tout cette attitude

Sur ce point précis, nous ne comprenons pas, là encore, l'obstination du Gouvernement, qui n'a rien de constructif ni de pragmatique Alors que Emmanuel Macron a fait campagne sur un discours très favorable aux entreprises, désignant même la simplification des obligations administratives qui pèse sur la vie des entreprises, notamment des plus petites, comme un volet prioritaire, voilà qu'il a fait le choix de reprendre une mesure mise en place par son prédécesseur, laquelle va représenter une charge notamment pour les plus petites entreprises, en termes de temps et de coût, évaluée

Nous ne comprenons vraiment pas ce choix. Nous proposons d'aider le Gouvernement en lui retirant cette épine du pied avec une solution alternative tout à fait viable, mais la main tendue est refusée. Où est donc ce « nouveau monde » promis par Emmanuel Macron ? Où est l'esprit constructif tellement vanté par la communication de La République En Marche ? Selon les Selon les audits commandés par Bercy à l'IGF, cette réforme devrait coûter entre 300 et 420 millions d'euros aux entreprises concernées, entre le paramétrage des logiciels, la formation des utilisateurs et la pédagogie à déployer auprès des salariés. Selon l'étude du cabinet Deloitte pour la délégation aux entreprises du Sénat, la facture pour les entreprises pourrait s'élever à 1,2 milliard d'euros la première année. Environ 75 % du coût total de la mesure reposera sur les très petites entreprises par l'effet de multiplication d'un coût fixe faible par un très grand nombre d'entreprises. La moitié du coût de la mesure correspondra au paiement des experts-comptables et des éditeurs de logiciels notamment. Ces prestataires de gestion de paye devraient en effet accroître le prix de leurs services rendus en raison des coûts de la mise en conformité de leurs outils. Pour eux, il s'agira vraiment d'un effet d'aubaine L'autre moitié du coût correspondra à un accroissement des coûts salariaux des entreprises. Cela est lié au temps supplémentaire consacré à communiquer auprès des salariés et à répondre aux différentes questions à la suite de la mise en oeuvre de la mesure. Cela comprend également la nécessité, dans certains cas, de demander un rescrit à l'administration fiscale pour confirmer le caractère imposable ou non de certains éléments de rémunération au titre de l'année de transition, sans compter les éléments de rémunération exceptionnels. Enfin, exceptionnels. Enfin, l'accroissement du temps de traitement des problèmes particuliers posés par les employés en situation de mobilité internationale doit Pour les entreprises se pose également le problème de l'engagement de la responsabilité juridique de l'entreprise. Un problème de plus, me direz-vous ! Au point où on en est ce n'est pas très grave. Dès lors que l'employeur devient le collecteur de l'impôt, il devient en même temps dépositaire du secret fiscal. Sa responsabilité pourrait également être mise en cause s'il n'appliquait pas le bon taux, s'il ne s'acquittait pas en temps et en heure de ses nouvelles obligations déclaratives, s'il ne respectait pas le délai de règlement ou l'obligation de confidentialité. Ce risque serait encore accru pour les entreprises embauchant des salariés en contrat à durée déterminée ou des saisonniers. Par ailleurs, de la perte de confidentialité pour les salariés ?

Demain, ce sont le chef d'entreprise et la direction des ressources humaines qui connaîtront le taux de l'impôt et les autres revenus éventuels du salarié, mais aussi de ceux du conjoint, ses revenus fonciers, ses revenus immobiliers, etc. Connues de la direction du personnel et des ressources humaines, ces informations pourraient avoir des conséquences néfastes lors des négociations salariales. Les principales victimes de la réforme pourraient être les femmes dont le conjoint perçoit une rémunération confortable. S'il est prévu la possibilité pour le salarié contribuable de rendre anonyme son impôt en recourant au taux forfaitaire neutre, ce choix pourrait néanmoins faire peser sur lui une sorte de suspicion. L'étude du cabinet Deloitte a fait part de cette très forte inquiétude des chefs d'entreprise, qui, pour 70 % d'entre eux, craignent une dégradation des relations sociales au sein de leur entreprise. Les employeurs craignent également de se retrouver impliqués dans le contentieux fiscal lié à la mise en oeuvre du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement

Les particuliers employeurs ne sauraient être assimilés à des entreprises. Leur moyenne d'âge, mis à part pour les gardes d'enfants, est de 65 ans. Beaucoup n'ont pas la maîtrise d'un ordinateur, ou ne résident pas dans une zone couverte par Internet. Des systèmes de chèques emploi service ont été conçus à leur intention. L'obligation, pour les intéressés, de prélever l'impôt sur le revenu à la source anéantirait la simplification ainsi réalisée. Le rapport d'audit de l'IGF a décrit les graves difficultés prévisibles. Notamment, le particulier employeur devrait déclarer le salaire de chaque mois huit à dix jours avant de l'avoir versé, alors que, le plus souvent, le nombre d'heures de travail effectuées durant ce mois n'est pas encore connu. De surcroît, les employeurs qui omettraient de verser au Trésor l'impôt retenu sur le salaire encourraient des sanctions. La crainte de celles-ci, de la part de personnes âgées mal équipées, ne peut qu'amplifier le recours au travail au noir. C'est d'ailleurs la conclusion de l'IGF. La solution proposée en première lecture par notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, que notre groupe Les Républicains tient à féliciter vivement pour le travail considérable qu'il a effectué sur ce sujet, permettrait de résoudre tous les problèmes exposés à l'instant. Mais le Gouvernement refuse de mettre à profit les résultats de ce travail pour trouver une solution qui soit acceptable et acceptée par tous. Dans ces conditions, le débat n'a plus lieu d'être prolongé, et c'est pour cette raison que le groupe Les Républicains votera la motion, déposée par la commission des finances, tendant à opposer la question préalable au second projet de loi de finances rectificative pour 2017. La discussion rectificative pour 2017. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

que les collectivités, puisque que vous parlez plus particulièrement d'elles, bénéficient- si l'on peut dire -d'un abaissement de la cotisation employeur maladie de 11,5 % à 9,9 %, tel que prévu par le décret examiné par le Conseil national d'évaluation des normes le 30 novembre dernier.

du Gouvernement est défavorable. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.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

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un processus législatif engagé avec la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Comme elle l'a fait dans un grand nombre de domaines, cette loi a habilité le Gouvernement- à l'époque contre l'avis du Sénat -à prendre par ordonnances des dispositions relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé. Le projet de loi dont l'adoption définitive est aujourd'hui soumise au vote de notre assemblée tend à ratifier l'une des deux ordonnances publiées sur ce fondement. Cette ordonnance, en date du 27 avril 2017, comporte des dispositions de nature et de portée très diverses. Plusieurs évolutions vont dans le bon sens, comme j'ai eu l'occasion de le souligner lors de l'examen en première lecture. Elles traduisent des recommandations formulées par le Conseil d'État ou la Cour des comptes, en réponse à certaines pratiques contestables relevées à l'occasion de contrôles ou de missions d'inspection, en assurant la conformité des instances disciplinaires aux exigences d'indépendance et d'impartialité ou encore en améliorant la transparence s'agissant de leur fonctionnement interne. Ces mesures contribueront à renforcer la nécessaire confiance des professionnels de santé à l'égard des instances ordinales. Pour autant, les évolutions apportées au texte du projet de loi, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, sont l'écho de questions soulevées par l'ordonnance et, sans doute, aussi, le signe d'une concertation insuffisante en amont avec les représentants des instances ordinales. Ceux-ci l'ont d'ailleurs regretté, alors même que plusieurs mesures auront des conséquences directes sur leur organisation et leur fonctionnement. Comme j'ai pu l'exprimer à cette tribune lors de l'examen en première lecture, la commission s'est interrogée sur la pertinence de certaines mesures, soit rigides, car imposant à tous des modes d'organisation plaidés par quelques-uns, soit susceptibles de faire peser sur les ordres des charges de gestion peut-être excessives. L'application aux conseils nationaux des règles en matière de marchés publics, en particulier, m'a semblé quelque peu disproportionnée alors même que certains ordres, comme celui des pharmaciens, se sont déjà engagés de leur propre chef dans une démarche de responsabilisation sur ces questions, ne serait-ce qu'au regard des comptes qu'ils doivent légitimement rendre à leurs membres. Si je comprends la finalité poursuivie par le Gouvernement, il nous faut aussi veiller à ne pas fixer des cadres trop rigides. Les positions adoptées par le Sénat en première lecture ont reflété ces réserves de notre commission des affaires sociales à l'égard de plusieurs dispositions de l'ordonnance. Après des échanges nourris avec le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire est néanmoins parvenue à un accord sur ce texte, qui reprend plusieurs apports du Sénat. La CMP a ainsi confirmé la suppression, sur l'initiative de notre commission, de la possibilité de remplacement des pharmaciens d'officine en cas de « circonstances exceptionnelles », formule aux contours jugés trop flous. On pouvait en effet s'interroger sur l'opportunité d'une nouvelle évolution, alors que la loi Santé a permis, encore récemment, une avancée pour tenir compte de situations individuelles. a également confirmé le maintien de la possibilité pour les membres en cours de mandat du conseil national d'être élus assesseurs à la chambre disciplinaire de l'ordre des pédicures-podologues. Notre souci, par cet ajustement, est de ne pas restreindre excessivement le vivier des « forces vives », en l'occurrence dans un ordre jeune, alors qu'existent par ailleurs d'autres règles permettant de respecter les exigences d'impartialité. D'un commun accord, nous avons supprimé, en outre, le caractère rétroactif de la présence de représentants de l'État au sein du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, afin d'éviter tout risque juridique. D'une manière plus générale, il nous est apparu important de stabiliser rapidement un texte afin de ne pas perturber le fonctionnement des instances ordinales en cours de renouvellement et de sécuriser leurs délibérations. C'est la raison pour laquelle il était important de parvenir en CMP à un accord sur ce texte. Dans cette finalité, nous avons notamment accepté de rétablir l'application aux conseils nationaux des ordres des principes et règles relatifs aux marchés publics, sous réserve toutefois d'une clarification adoptée sur mon initiative. Il ne saurait en effet être question d'appliquer aux ordres, qui ne sont pas financés par des fonds publics, des règles de procédures plus strictes que celles qui sont valables pour les administrations en deçà d'un certain seuil, la mise en concurrence ne devra donc pas être obligatoire. Madame la ministre, ces dispositions s'appliqueront à compter de 2020, dans des conditions et sous réserve d'adaptations prévues par décret. Je souhaite que ce temps de préparation soit mis à profit par vos services pour engager un dialogue serein avec les représentants des ordres des professions de santé et, ainsi, ajuster les règles de droit commun complexes à leurs besoins réels, selon une approche pragmatique. Nous resterons vigilants à ce sujet. Au nom de la commission des affaires sociales, je vous invite, mes chers collègues, à adopter ce projet de loi de ratification d'ordonnance, dans le texte équilibré tel qu'issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

a pour objectif de renforcer l'indépendance et l'impartialité des juridictions ordinales, ainsi que de faire évoluer les compétences des organes des ordres et permettre l'application par leurs conseils nationaux de la législation ayant trait aux marchés publics. Cette ordonnance comporte un certain nombre de recommandations issues du Conseil d'État- précisément de la Mission d'inspection des juridictions administratives -, de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des affaires sociales- -qui ont successivement conduit depuis 2012 des missions d'inspection et de contrôle portant sur les ordres des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des masseurs-kinésithérapeutes. Cette ordonnance comporte trois chapitres, qui concernent le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et, enfin, les dispositions transitoires et finales. Je me félicite qu'un accord ait été trouvé en commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le 5 décembre dernier. Les accords ont notamment supprimé l'article 3 , qui tendait à interdire le cumul entre fonctions d'assesseur d'une instance disciplinaire et fonctions de président et secrétaire général de l'organe de l'Ordre. La CMP a également réécrit l'article 4, introduit par un amendement gouvernemental au Sénat. Cette modification permet d'organiser la présence des représentants du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de la santé aux délibérations du Conseil national de l'ordre des pharmaciens pour l'avenir, et non de façon rétroactive à compter d'avril 2017. Enfin, la CMP n'a pas retenu l'article 4 , visant à supprimer l'extension aux conseils nationaux des ordres des grands principes des marchés publics. Cela a permis de modifier le texte pour en faciliter l'appropriation par les ordres, qui sont conduits à l'appliquer, sans pour autant dénaturer les objectifs structurels que Le projet de loi, qui comportait initialement un seul article, en compte dorénavant dix. Il prévoit ainsi un certain nombre de dispositions applicables, sans distinction, à tous les ordres. Je souligne que, pour permettre aux ordres de s'adapter au nouvel environnement juridique, certaines mesures feront l'objet d'une application progressive, notamment le renouvellement des instances ordinales, la certification des comptes combinés et l'application des règles de marchés publics. Pour finir, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier Mme la rapporteur Corinne Imbert pour son rôle dans la recherche d'une solution consensuelle et la qualité des échanges. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis pour le vote des conclusions de la CMP sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé, en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et sur recommandation du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de l'IGAS. Le rapport 2017 de la Cour des comptes a émis un avis sévère à l'encontre de l'ordre national des chirurgiens-dentistes défaut de représentativité et de renouvellement des instances dirigeantes, absence de contrôle sur son mode de fonctionnement, défense d'intérêts catégoriels qui ne lui incombe pas, ou encore désordres graves dans les comptes et la gestion. La Cour des comptes, qui rappelle à cette occasion la mission de service public de l'ordre des chirurgiens-dentistes, invite le législateur à introduire davantage de transparence, d'indépendance et d'impartialité dans les conseils nationaux des ordres des professions de santé. Sur ces trois points, nous ne pouvons que saluer les améliorations proposées dans cette ordonnance. Nous saluons ainsi l'accord trouvé en commission mixte paritaire et le dialogue mené par les deux rapporteurs, en bonne intelligence. Ce travail a permis l'élaboration d'un texte enfin stabilisé. Nous regrettons toutefois les conditions de concertation, qui n'ont pas été jugées satisfaisantes par les ordres et qui ont conduit à l'introduction de plusieurs articles supplémentaires lors de l'examen du texte par le Parlement. Des concertations plus poussées en amont auraient pu permettre l'émergence d'un texte certainement plus consensuel dès le départ. Comme l'a indiqué en première lecture mon collègue Guillaume Arnell, nous sommes bien conscients de la lourdeur des procédures et des surcoûts induits par le besoin de transparence. S'agissant des règles des marchés publics, certains ordres les appliquent déjà ; il convenait d'adapter ces dispositions par un texte réglementaire. nationale et le Sénat ont toutefois écouté les remarques des professionnels, notamment en reportant à 2020 l'application des règles de marchés publics et de certification des comptes, afin de permettre aux ordres de s'y préparer. La CMP a également permis d'assurer que les ordres, qui sont bien sûr financés par de l'argent privé, ne se voient pas appliquer des dispositions plus contraignantes que celles qui concernent les administrations ou les établissements publics. Cette rédaction nous semble raisonnable et acceptable par tous. de l'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur d'une instance disciplinaire et les fonctions de président ou secrétaire général d'un conseil de l'Ordre, il apparaît effectivement nécessaire d'éviter les confusions entre les autorités de poursuite et les autorités de jugement, comme l'a souligné le rapporteur de l'Assemblée nationale, que je rejoins sur ce point. De même, nous pensons que les avancées en matière de règlements intérieurs sont absolument nécessaires, et nous sommes satisfaits de l'accord trouvé. Le groupe du RDSE votera donc en faveur du texte élaboré en CMP par les deux assemblées.

Je salue l'aboutissement de la CMP et me réjouis de pouvoir discuter d'un texte qui, au travers d'un équilibre certain, permettra aux différents ordres d'évoluer avec un cadre juridique plus solide. Oui, ce texte est une bonne nouvelle, et une avancée certaine que le législateur et professionnel de santé que je suis applaudit. L'ordonnance en question modifie plusieurs codes- vous les avez rappelés, madame la ministre : le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique -afin de permettre aux ordres un fonctionnement optimisé et garantir leur indépendance. Elle modifie aussi leurs conditions de gestion par la réforme de la certification des comptes, l'application des règles de marchés publics et la généralisation d'un règlement intérieur.

il apparaissait nécessaire d'encadrer au mieux les conditions d'exercice des membres de ces ordres. Oui, mes chers collègues, la défiance ambiante touche toutes les institutions et, admettons-le, les critiques sur la gestion parfois opaque des ordres n'ont pas toujours été infondées. Je suis donc satisfait de la mise en place d'une gestion financière plus transparente, qu'elle concerne la certification des comptes ou la passation des marchés. l'évolution des compétences des organes, l'ordonnance réaffirme l'importance des échelons régionaux des ordres des professions de santé, en leur donnant une plus grande latitude en matière d'organisation et en renforçant leur rôle en matière budgétaire.

Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Il est essentiel que la population et les professionnels de santé aient confiance dans l'organisation des ordres au niveau tant régional que national, dans leur gestion patrimoniale et dans l'impartialité de leurs instances juridictionnelles. Enfin, madame la ministre, je salue, en plus de la volonté de concertation avec les principaux intéressés, le souhait pratique d'une application progressive de certaines mesures, afin d'assurer une transition pérenne pour le renouvellement des instances ordinales, les nouvelles modalités de passation de marchés publics ou de certification des comptes, en laissant le temps aux ordres de s'approprier le nouveau cadre de leur exercice. Le groupe La République En Marche soutient cette démarche très pragmatique et votera le texte de ratification. Il suivra aussi avec attention les décrets d'application de ce dernier.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, n'est-il pas paradoxal, pour un gouvernement qui prétend représenter le nouveau monde, de soumettre une ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé qui semble dater d'un autre temps, d'autant que ces ordres ne font pas l'unanimité ? Ainsi, le 12 mai 2016, la promulgation du code de déontologie des infirmiers a été retoquée par l'Autorité de la concurrence, au motif que « l'approche retenue par l'ONI [l'Ordre national des infirmiers] paraît particulièrement préjudiciable à la profession d'infirmier ». Répondant à une question posée à l'Assemblée nationale en août 2016, Marisol Touraine, alors ministre des affaires reconnaissait que seulement 177 000 des 640 000 infirmiers avaient adhéré à l'Ordre, ces chiffres intégrant les 15 % d'infirmiers diplômés d'État libéraux obligés de cotiser pour être remboursés par la sécurité sociale ! On est loin d'une adhésion massive de la profession. D'ailleurs, toutes les professions de santé ne sont pas régies par un ordre : je pense à la profession d'orthophoniste, qui n'a pas d'ordre et fonctionne parfaitement ! C'est vrai ! Créés voilà dix ans, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les ordres professionnels se sont vu confier des missions auparavant dévolues aux structures publiques, comme l'enregistrement et la gestion des tableaux de démographie des professions en déterminant les besoins en formation selon la population.

ne se fonde le plus souvent que sur la menace de sanctions. Devant le danger de voir encourager le corporatisme et la rivalité avec les autres professions, plutôt que de supprimer les ordres professionnels ou, du moins, de rendre facultatives leurs adhésions, quelles modifications votre gouvernement souhaite-t-il apporter, suite des dysfonctionnements relevés par l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, le Conseil d'État et la Cour des comptes, l'ordonnance modifie les règles de composition et d'élection des conseils des ordres. Elle vise également à consolider les règles de gestion interne et à renforcer l'impartialité des instances disciplinaires. Le renforcement de la régionalisation de la santé, avec la réforme territoriale, entraîne l'adaptation de l'organisation des échelons territoriaux des ordres professionnels, ce que prend en compte cette ordonnance. Elle étend ainsi à l'ensemble des conseils nationaux et régionaux des ordres la possibilité pour leur président d'agir en justice, alors que cette faculté était prévue jusqu'à présent L'ordonnance modifie également la composition des conseils, la répartition des sièges au sein des différents échelons et les modes d'élection et de désignation, de manière à simplifier les règles et à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l'ensemble des conseils. Si cette mesure est positive, nous ne pouvons que regretter le fait que le Conseil national de l'Ordre demeure exclu de l'obligation de parité. Enfin, cette ordonnance renforce le contrôle des ordres sur les avantages consentis aux professionnels de santé par des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé. Cela fait suite au scandale du Mediator. Désormais, les professionnels de santé doivent rendre publics leurs liens avec les entreprises de produits de santé. Les montants des conventions signées entre les acteurs du système de santé et les industriels devront être publiés à partir d'un seuil de dix euros, sur un portail dédié. Il revient ainsi à chaque citoyenne et citoyen de connaître en toute objectivité la nature des relations qui lient les industries de santé aux professionnels de santé. Cette ordonnance apporte donc de petites améliorations au fonctionnement interne des ordres professionnels, mais ne règle aucunement le problème, à savoir l'existence même des ordres professionnels. Plusieurs ministres de la santé de gouvernements de couleur politique différente avaient reconnu la nécessité de remettre en question ceux-ci, mais ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. Pour quelles raisons ? Ne s'agit-il pas du poids des intérêts en cause ? Les ordres sont, dans les faits, des acteurs sensibles aux politiques de maîtrise des dépenses de santé, voire des facilitateurs. Ceci explique sans doute cela Faire porter sur l'individu la responsabilité des manquements à la déontologie sans prendre en compte les conditions d'exercice qui sont imposées aux personnels soignants par le vote de budgets toujours plus indigents est bien pratique. Et pourquoi faudrait-il payer en adhérant à une instance ordinale pour, tout simplement, exercer son métier ? Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, mon groupe votera contre ce texte. Nous appelons de tous nos voeux le vote d'un décret qui supprime les ordres. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues,

Il nous a fallu, pour aboutir, faire certaines concessions. Je tiens d'ailleurs à remercier ma collègue et rapporteur, Corinne Imbert, d'avoir trouvé un consensus avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Il nous semblait utile que les règles applicables à ces ordres soient revues, afin d'en garantir la fiabilité. Les recommandations du Conseil d'État, de l'IGAS et de la Cour des comptes formulées à ce titre se retrouvent donc dans ce texte. Il fallait en effet renforcer les règles en matière de transparence, ainsi que les exigences d'indépendance et d'impartialité des instances disciplinaires. Cela passait par conséquent par la définition de dispositions communes les concernant. Le Sénat a ainsi concédé le maintien de l'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur d'une instance disciplinaire et celles de président ou de secrétaire général du conseil de l'ordre. Il a concédé également le maintien de l'obligation, pour les conseils nationaux des ordres, d'élaborer un règlement intérieur. Nous avions supprimé cette disposition, car certains ordres disposent déjà d'un tel règlement. Le Sénat a enfin concédé l'application aux ordres des règles en matière de marchés publics, tout en adoptant une clarification- comme l'a souligné Mme la rapporteur -, afin de s'assurer que les ordres ne se voient pas appliquer des dispositions

mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur l'un des projets de loi de ratification d'ordonnances rédigées en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, votée sur l'initiative de la précédente ministre de la santé, Marisol Touraine, que nous avions soutenue dans sa démarche. L'attitude du groupe socialiste et républicain s'inscrit aujourd'hui dans le prolongement de ce positionnement. L'ordonnance relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé renforce l'indépendance et l'impartialité des juridictions ordinales,

Elle prend en compte les diverses recommandations formulées et les dérives dénoncées tant par le Conseil d'État que par la Cour des comptes, ou encore par l'Inspection générale des affaires sociales, dans le cadre de leurs missions d'inspection et de contrôle portant sur différents ordres. La mesure visant à rendre applicables aux conseils nationaux les grands principes des marchés publics avait suscité, dans un premier temps, certaines réticences. Pour autant, l'application des grands principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ne nous paraît pas discutable. cette mesure en première lecture, le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire nous semble satisfaisant. Les ordres ont une mission de service public, mais ne sont pas financés par des deniers publics. Aussi, si des règles de transparence s'imposent, elles ne sauraient être plus plus contraignantes que celles qui sont applicables aux organismes publics. La rédaction qui permet aux ordres d'organiser des procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalable en deçà de certains seuils, en fonction de leur objet ou de leur valeur estimée, nous paraît aboutir à une conciliation bienvenue entre la responsabilisation des ordres et les exigences de transparence et de mise en concurrence. Le groupe socialiste et républicain votera donc ce texte, qui maintient la cohérence de notre système de santé sans l'accabler de règles obscures et alambiquées ni l'amputer imprudemment de tout encadrement. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions professions de santé est un sujet extrêmement sensible. Est-il ainsi besoin de rappeler que la commission des affaires sociales s'était opposée à cette habilitation en critiquant l'illisibilité des mesures proposées, lors de son premier examen, en octobre 2017 ? Cela me semble être un signal d'alerte important, nous invitant à la plus grande prudence dans nos débats.

et l'ordonnance d'avril 2017, visant le projet de loi de ratification. Le Gouvernement avait alors justifié ce choix pour des raisons de sécurité juridique. Le nouveau projet de loi nous paraît beaucoup plus clair et équilibré de ce point de vue. En effet, les services de l'État ont procédé à plusieurs correctifs pour assurer une cohérence globale de ce texte : évolution de la composition et des compétences des organes composant les ordres, allégement des procédures, renforcement des moyens destinés à veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis par les entreprises, modalités d'intervention des ordres en matière d'exercice professionnel, etc. Ces ordonnances assurent donc une plus grande indépendance de la profession et une amélioration de sa gestion. En bref, cette ordonnance du 27 avril 2017 semble une mesure de bon sens et recueille tout l'assentiment de mon groupe. Elle améliore en effet la transparence dans le fonctionnement interne des ordres. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, ou encore l'IGAS ont relevé de nombreuses fois les dysfonctionnements des ordres des professions de santé, notamment ceux de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Les modifications relatives à l'amélioration de la gestion de la situation patrimoniale et financière, à l'application des règles des marchés publics, ou encore la mise en place de règlements publics sont plus que vertueuses. En outre, ces ordonnances mettent les instances disciplinaires en conformité avec les exigences d'indépendance et d'impartialité. En appliquant aux conseils nationaux les principes et procédures des marchés publics, le Gouvernement veut moderniser ces instances : édiction d'un règlement intérieur, publication d'un rapport d'activité, certification des comptes combinés, responsabilité du suivi de la politique immobilière, etc. Cette nouvelle transparence des ordres des professions de santé est donc salutaire. Néanmoins, l'absence de concertation avec les sept ordres professionnels est dommageable à cette ordonnance. Des recours ont ainsi été déposés devant le juge administratif, alors que ce texte vise à assurer une activité plus utile et pertinente de ces institutions. Il faut que la refonte des organisations des ordres concoure à une rationalisation des systèmes en place, en fusionnant des conseils des ordres, et à une réforme des instances disciplinaires, permettant aux professionnels de santé d'être jugés par leurs pairs. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, mon groupe votera le texte établi par la commission mixte paritaire. Celui-ci propose un équilibre raisonnable et nous paraît aller dans le sens d'une modernisation vitale de notre système de santé. La

nous arrivons à l'ultime étape de la navette pour ce projet de loi qui prévoit la ratification de l'ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé. Je tiens, tout d'abord, à féliciter ma collègue rapporteur, Corinne Imbert, pour la qualité de son travail qui a notamment permis à la commission mixte paritaire d'aboutir à un accord.

Le projet de loi que nous examinons modifie le fonctionnement des ordres. D'une part, il vise à renforcer les conseils nationaux en leur donnant la possibilité d'ester en justice ou de se porter partie civile. D'autre part, il modifie leurs conditions de gestion en prévoyant plusieurs mesures, comme la certification des comptes combinés au niveau national, l'application des règles relatives aux marchés publics, la généralisation d'un règlement intérieur. L'ordonnance tend également à préserver l'indépendance et l'impartialité des ordres et de leurs juridictions avec la mise en place d'un régime d'incompatibilité et d'un encadrement du régime indemnitaire. En première lecture, nous avons soutenu les mesures qui améliorent la transparence interne de ces instances ou qui renforcent les exigences d'impartialité. Elles vont dans le bon sens et doivent consolider la nécessaire confiance des professionnels de santé à leur égard. Néanmoins, le Sénat s'était interrogé sur la pertinence de certaines évolutions, susceptibles de faire peser sur les ordres de lourdes charges de gestion. Le travail et l'écoute des rapporteurs de chacune des assemblées nous permettent de nous prononcer aujourd'hui sur un texte équilibré, conservant des apports du Sénat qui ont été clairement présentés par Corinne Imbert. Je n'y reviens donc pas. Le groupe Les Républicains votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire, afin de permettre l'application rapide de ce texte pour ne pas perturber le fonctionnement des instances ordinales en cours de renouvellement. La discussion

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

adopté cette posture ? Nous avions la volonté de donner la possibilité aux départements, mais également aux régions- c'est l'une des dispositions que le Sénat a permis d'adopter -de continuer à intervenir dans le domaine de la GEMAPI au-delà de 2020.

et syndicats mixtes, avec la faculté de ne transférer qu'une partie de leur compétence, voire une partie de chacune des quatre missions constitutives de cette compétence, à un ou plusieurs syndicats sur tout ou partie de leur territoire.

d'adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, tel qu'un établissement public territorial de bassin. Nous avons voulu également permettre un régime transitoire de responsabilité des communes

fut très bref dans un domaine éminemment technique. Mais nous avons souhaité aller de l'avant et permettre à ce texte d'aboutir, car il est utile que les intercommunalités disposent des diverses possibilités de transfert et de délégation décrites ci-dessus dès leur prise de compétence au 1 janvier 2018, afin de ne pas retarder les délibérations. Enfin, il est bon que le régime de responsabilité

les communes isolées ne sont pas oubliées, qu'il s'agisse du régime de responsabilité limitée ou des conventions passées avec les départements ou avec les régions.

Le vote de ces conclusions constitue, au surplus, l'aboutissement législatif, atteint en l'espace de deux mois, de l'un des chantiers lancés au sein de la Conférence nationale des territoires : deux mois, c'est rapide, et je sais l'énergie et l'engagement dont ont fait preuve

Vous le savez, le Gouvernement, attentif aux préoccupations exprimées par les territoires et leurs élus locaux, a fait le choix de la stabilité. L'équilibre en matière de répartition des compétences, qui résulte notamment des lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015, doit désormais s'appliquer.

qui sont intimement liées, ainsi que leur transfert à l'échelon intercommunal à compter du 1 janvier 2018, constituait une avancée importante de la loi du MAPTAM du 27 janvier 2014. De ce point de vue, la GEMAPI a suivi une logique forte, une logique de solidarité. Toutefois,

Il permet aux départements de continuer à défendre les stratégies et les politiques qu'ils ont su mettre au point ; il étend cette faculté aux régions, qui exercent des attributions en ce domaine et qui souhaitent il affirme clairement un principe de sécabilité des différentes composantes de la compétence GEMAPI qui seul garantit aux collectivités territoriales leur libre organisation dans l'exercice de cette compétence ; il crée un régime de responsabilité adapté aux transferts d'ouvrages aux intercommunalités,

Ce compromis était important pour la clarté de l'exercice de la compétence GEMAPI, à un peu plus de dix jours de son transfert aux EPCI : je me félicite que les réserves exprimées par le Gouvernement sur ce point aient été entendues.

C'est pourquoi, en remerciant de nouveau le Sénat de sa contribution active et positive à ce débat, le Gouvernement ne peut que vous appeler à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire qui vous sont soumises. La parole

territoriale nouveau et, reconnaissons-le, partiellement inachevé. Je fais partie de la vaste majorité qui, au Sénat, a adopté la loi NOTRe. au terme d'un compromis laborieux, pour lequel tout le monde a dû faire quelques efforts, ce texte comportait cet objet nouveau : la définition de la compétence relative aux milieux aquatiques et à la protection des inondations.

des attentes, mais aussi un peu d'incompréhension et, disons-le, certaines préventions dans cet hémicycle. Quand je me souviens de l'état d'esprit dans lequel nous avons discuté avec de nombreux membres du Parlement

Étant commis à d'autres missions en rapport avec ce qui se passe au sein de la Conférence des territoires, j'ai, pour ma part, la conviction que ce travail s'approfondira encore dans les mois à venir.

on garantit une plus grande souplesse d'exécution en permettant de recourir aux outils institutionnels locaux déjà éprouvés, que ce soit vers le plus haut,

article énonce qu'une collectivité territoriale peut déléguer à une autre collectivité d'une autre catégorie toute compétence dont elle est attributaire. Je suis frappé de constater

des objets techniques, se trouve un autre sujet : le financement de la compétence. Selon moi, l'assise de la compétence GEMAPI sur un impôt direct ajouté aux prélèvements existants n'est ni complètement rationnelle ni complètement équitable. Dans un autre exercice, nous serons appelés, avec tout un collège

des débats que nous avons consacrés, au sein de la Haute Assemblée, à ce sujet extrêmement important. La présente proposition de loi vient assouplir, fort heureusement,

faute d'étude d'impact préalable. Force est de constater aujourd'hui que ces dispositions sont inopérantes. À quelques jours du transfert programmé au bloc local,

alors même que cette expertise eût été nécessaire pour légiférer correctement. Je pense notamment à la maîtrise des eaux fluviales et au ruissellement, qui, peut-on dire, ont fait l'objet d'un compromis : à ce sujet, on a renvoyé à la réalisation d'un rapport par le Gouvernement.

Les élus n'auront d'autre solution que de choisir entre deux contrariétés : imposer à leurs administrés une nouvelle taxe ou amputer leur budget. Pour ceux qui vont créer ce nouvel impôt assis en partie sur la taxe d'habitation, le manque de visibilité à court terme est fâcheux.

de loi de finances. Ces instances accompagnent les collectivités territoriales dans la prise de compétence GEMAPI et soutiennent leurs actions par le biais de la réalisation d'études et de travaux. étant, ne boudons pas notre plaisir : la proposition de loi GEMAPI va dans le bon sens. Elle corrige l'infaisable. Elle fait confiance à l'intelligence territoriale assouplit des dispositions que le bloc communal aurait été dans l'incapacité de mettre en oeuvre. À ce titre, je salue la volonté du Gouvernement, la sagesse du Parlement, tout particulièrement celle du Sénat, et l'excellent travail accompli par notre rapporteur, ... C'est bien rapidement, même si ce n'est que de manière incomplète. Nous devrons nécessairement nous revoir pour légiférer de nouveau, et cette fois, je le souhaite, de manière pérenne et stable, au titre de cette compétence.

a été rappelé au cours de nos différents échanges : la compétence GEMAPI permet de répondre aux défaillances révélées par différents phénomènes climatiques qui ont causé des pertes humaines

Toutefois, nous l'avons rappelé précédemment, la mise en oeuvre de cette compétence est techniquement complexe : elle le reste. Sa structuration institutionnelle est difficile et le partage des responsabilités est toujours flou.

Cette proposition de loi clarifie et assouplit une partie du dispositif et rassure les élus locaux en raison de la pérennisation des engagements pris par les régions et les départements, de l'extension de l'assistance technique des départements

et en débattre : il était plus que contraint, voire de l'ordre de l'urgence, et ce n'est pas sans conséquence, alors même que les enjeux en termes de sécurité pour les personnes et les biens sont centraux. De nombreux travaux ont porté sur les contraintes temporelles qui pèsent sur les travaux parlementaires, et nous en avons de nouveau une illustration ici. à force de pallier les difficultés d'un texte qui est nécessaire dans sa thématique, mais insuffisant dans ses modalités, on risque de créer d'autres difficultés

Ensuite, cela a été souligné, mais j'y insiste, il est évident que des problèmes essentiels ont été négligés. Je ne reviendrai pas sur l'absence de traitement des grands corridors fluviaux, ni sur la problématique spécifique des territoires littoraux,

Malgré ces insuffisances, cette proposition de loi répond pour partie, je l'ai dit, aux interrogations opérationnelles des élus locaux, tout en restant malheureusement, si vous me permettez l'expression, au milieu du gué. Nous formulons par ailleurs le voeu que les différents rapports que le Gouvernement remettra au Parlement couvrent l'ensemble des problématiques évoquées précédemment et puissent- enfin ! -faire l'objet d'un véritable temps de réflexion et d'expertise de la part du Sénat. Bref, Bref, au final, pour reprendre une image de saison- nous nous rapprochons de Noël -, mieux vaut se rassurer en se disant qu'il est préférable d'avoir une part de dinde que pas de dinde du tout ! Très bien ! Cela étant, vu mon département d'élection, je vous recommande le canard

La commission mixte paritaire a su conserver l'esprit de ce texte. Assouplir sans faillir : cela aurait pu être le mot d'ordre de cette proposition de loi, déposée par le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés à l'Assemblée nationale, qui vise- il est utile de le rappeler -à permettre aux départements et à leurs groupements de continuer à exercer la compétence GEMAPI jusqu'au 1 janvier 2020. C'est un effort d'écoute du terrain et de considération des élus, auquel mon groupe, Les Indépendants-République Un certain nombre de mesures avaient déjà été prises pour faciliter le transfert des compétences de l'eau. Le travail des missions d'appui technique de bassin mérite, de ce point de vue, d'être salué. D'ailleurs, un amendement déposé à l'Assemblée nationale, en séance publique, visait à prolonger ce travail jusqu'en 2020. Notre chambre n'a finalement pas retenu

d'affecter une partie de la taxe GEMAPI au paiement des dépenses relatives à la protection contre les inondations ou les coulées d'eaux boueuses après orage. Cette disposition est essentielle pour protéger nos populations. En effet, les départements connaissent de vraies difficultés financières, vous le savez comme moi, mes chers collègues, dans l'exercice de ces missions. La CMP n'a pas, non plus, retenu l'article 9, introduit en séance publique, lundi dernier, par le Sénat. La mesure qu'il comportait permettait pourtant, elle aussi, de lutter contre un autre problème de taille : le ruissellement des eaux pluviales. En affectant une partie de la taxe GEMAPI à l'exercice de ces missions, la proposition de loi prenait à bras-le-corps cette problématique et mettait en place un dispositif d'accompagnement financier des collectivités territoriales. Députés et sénateurs ont en revanche trouvé un compromis dans la nouvelle rédaction de l'article 5 : la proposition d'un rapport sur la répartition des compétences GEMAPI entre collectivités et groupements, la clarification de l'articulation entre mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et celle de lutte contre l'érosion des sols et l'amélioration du financement des opérations et équipements affectés à ces missions sont trois enjeux de taille. Le groupe Les Indépendants-République et Territoires approuve la prise en compte de ces enjeux.

Si nous regrettons que ce dernier n'aille pas suffisamment loin dans la transformation de notre modèle GEMAPI- nous y reviendrons, je le sais -, il pose la première pierre d'un édifice à construire et apporte une souplesse nécessaire aux collectivités dans l'évolution de leurs compétences. La

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il me revient la responsabilité de clôturer la discussion générale d'un texte examiné au pas de charge. Je ne reviendrai pas sur les réserves exprimées, en première lecture ni sur la méthode qui a présidé à l'examen de ce texte. À ce titre, je veux saluer le travail du rapporteur, Mathieu Darnaud, fin connaisseur de ces problématiques et qui a su oeuvrer, avec talent, dans l'urgence. Le texte issu de nos travaux assume son ambition limitée : corriger quelques imperfections, sans bouleverser de nouveau l'organisation des territoires ni revenir sur l'esprit qui a entouré la création de la GEMAPI. Cette dernière a pour vertu de clarifier la gouvernance et de mieux coordonner les interventions entre les différents acteurs. Il importe donc que les aménagements que nous lui apportons ne constituent pas un détricotage ou un retour à la situation antérieure, qui a démontré ses failles et insuffisances. Parmi les éléments de souplesse apportés, je voudrais tout d'abord évoquer la sécabilité du transfert et de délégation de tout ou partie de la compétence GEMAPI, inscrite à l'article 3, au profit des syndicats, C'était une demande forte des élus. Le texte définitif prévoit toujours que les départements et les régions qui exercent cette compétence pourront continuer à le faire après 2020. En cette matière, la conclusion d'une convention quinquennale doit permettre de déterminer « qui fait quoi » et « qui paie quoi Les régions pourront aussi contribuer au financement de projets relevant de la GEMAPI et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte. En matière de responsabilité, les inquiétudes des élus étaient fortes. Le régime de responsabilité limitée, tel que nos travaux l'ont fixé, est de nature à lever certaines appréhensions. Je me réjouis aussi du compromis trouvé en CMP sur la question de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement qui a fait l'objet d'intéressants échanges en première lecture. La demande de rapport dans un délai de deux mois permet de la maintenir à l'agenda politique et parlementaire et d'évaluer au mieux les conséquences d'un transfert qui sera loin d'être neutre sur le plan financier pour nos nouvelles intercommunalités déjà chahutées. Par ailleurs, nous nous réjouissons que l'amendement soutenu par notre collègue Stéphane Artano et adopté par notre assemblée ait été repris dans le texte issu des

Je pense notamment aux îles maritimes composées d'une seule commune, qui sont, par nature, exposées au risque de submersion marine, mais qui ne disposent pas des moyens financiers ni de l'ingénierie pour assurer cette compétence. D'une manière générale, les conclusions de ce rapport d'évaluation seront donc, vous l'aurez compris, particulièrement attendues. Lors de la discussion générale de ce texte en première lecture, j'avais partagé mon expérience d'élue d'un massif, les Pyrénées, où les inondations peuvent être d'une grande violence, dans une version torrentielle où le transport solide est bien plus souvent dévastateur que le débit liquide. Je souhaite aussi attirer votre attention sur des territoires aux contraintes différentes : les anciens bassins miniers, chers à nos collègues Jean-Pierre Corbisez et Véronique Guillotin, profondément oubliés dans la version initiale de la GEMAPI. Très bien ! Ils se caractérisent par des sous-sols percés de nombreuses galeries, dont la plupart ont été noyées à la fin de l'exploitation minière. Le phénomène de remontée des eaux de nappe, observé depuis lors, porte des risques réels d'inondations. Le transfert de la compétence GEMAPI ne saurait exonérer l'État et les Charbonnages de France de leur responsabilité de réparer les stigmates de l'activité minière. Je vous rappelle qu'il existe déjà des contentieux, notamment en raison de l'affaissement de certains terrains. Les élus de ces anciens bassins miniers souhaitent donc obtenir la garantie que leur responsabilité ne sera pas engagée pour des inondations liées aux mines qui ont été exploitées sur leur territoire. D'autres lacunes que nous avons relevées lors de l'examen en première lecture n'ont évidemment pas été comblées. Je pense notamment aux questions relatives au trait de côte et à l'érosion marine. Le réchauffement climatique aura pour conséquence- c'est déjà le cas -une montée du niveau des océans et un renforcement des aléas climatiques. L'examen d'une proposition de loi de notre collègue Michel Vaspart nous donnera l'occasion, je l'espère, d'aborder ces thématiques dès le mois de janvier prochain. aussi de m'attarder sur une autre des ellipses de ce texte : la question du financement de la GEMAPI. Eh oui ! Disons-le d'emblée, l'État ne peut se décharger sur les collectivités territoriales de responsabilités nationales. À cet égard, les programmes d'actions de prévention des inondations- les fameux PAPI -devront continuer à soutenir la prise de compétence de la GEMAPI de façon importante par le biais des fonds Barnier. En effet, si la GEMAPI apporte cohérence et clarification, le transfert de charges afférent n'est pas anodin pour les collectivités, car nous savons le coût des ouvrages concourant à la GEMAPI. Si j'osais, je soulignerais aussi les difficultés réglementaires auxquelles les élus devront faire face, confrontés à une loi sur l'eau fréquemment inadaptée à certaines typologies de cours d'eau des procédures longues, trop longues, coûteuses et bien souvent mal appropriées, notamment dans les territoires de montagne. En dépit des réserves que j'ai formulées, cette proposition de loi tient compte de la diversité des territoires, car, comme je viens de l'évoquer, les problématiques ne sont pas les mêmes à Oignies, dans le Pas-de-Calais, à Miquelon-Langlade, ou chez moi, dans la vallée des Gaves. En un mot, ce texte donne aux collectivités plus de latitude pour s'organiser et fait davantage confiance à l'intelligence territoriale.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Personne ne demande la parole ?